Monsieur le président, La séance est reprise. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

dont une relative à la formation des ministres du culte, adoptée par charité, la majeure partie du texte ayant été vidée de sa substance. Nous n'avons eu de cesse d'alerter.

J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

en dehors du fléchage, dans les métropoles. Le texte dont nous débattons vise à remettre les communes au coeur de l'action intercommunale,

Nous souhaitons, par cet amendement, donner la possibilité aux adjoints des communes membres d'une intercommunalité de siéger dans les commissions intercommunales liées au sujet dont ils ont la charge dans leur commune, même lorsqu'ils ne sont pas conseillers communautaires. Cette possibilité répond à une demande largement répandue chez les élus locaux, qui ont trop souvent le sentiment que les intercommunalités se sont substituées aux communes. Je crois que nous partageons tous le constat que ce sentiment, malheureusement fondé, traduit une dérive par rapport à la fonction première des intercommunalités. Un aspect de ce problème général irrite tout particulièrement les élus municipaux : l'impression de ne plus savoir ce qui se décide dans leur territoire et de ne plus avoir voix au chapitre. Autoriser les adjoints des communes et les conseillers municipaux délégués à siéger dans les commissions intercommunales garantirait aux élus municipaux la possibilité de suivre les dossiers du territoire de l'intercommunalité concernant directement les sujets dont ils ont la charge. De cette façon, on réduirait le sentiment qu'ont les adjoints municipaux d'être tenus à l'écart d'un territoire dont ils sont pourtant les premiers élus. Les commissions intercommunales n'ayant pas de pouvoir décisionnaire, la question de la représentativité ne fait, à notre sens, pas obstacle à cette proposition. Il s'agit simplement d'offrir la possibilité à tous les élus municipaux intéressés de suivre les dossiers qui les concernent et de faire profiter l'intercommunalité de leur expérience et de leur connaissance du terrain, au travers des recommandations que ces commissions produisent. Une telle modification nous semble relever de la nécessité si l'on souhaite redonner aux communes la place qu'elles n'auraient jamais dû perdre. En garantissant aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués d'être intégrés à part entière dans le travail effectué par l'intercommunalité, on affirme que celle-ci a vocation à travailler avec les communes, et non à les remplacer. Quel

aux commissions intercommunales. Cette avancée importante me semble répondre à votre demande. En outre, il appartient à chaque EPCI, dans le cadre du pacte de gouvernance,

communautaire. Ainsi, dans tous les cas, la commune a la garantie d'être toujours représentée, ce qui permet notamment aux maires qui siègent au bureau communautaire, parfois d'ailleurs comme seul représentant de leur commune, d'être représentés dans cette instance qui est importante dans la vie communautaire. Quel est l'avis de la commission

et inscrire dans la loi que l'on permet à des conseillers municipaux d'y assister, alors que ces réunions ne sont pas ouvertes aux conseillers communautaires,

pour plus d'une réunion, par un conseiller municipal de leur commune. Il s'agit d'encourager les liens entre l'EPCI et la commune, en donnant plus de flexibilité au dispositif actuel de l'article 3.

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une partie- j'insiste sur ce point -d'une proposition de loi que j'avais déposée avec le groupe socialiste et républicain et qui a été adoptée par le Sénat. Il s'agit de mettre en oeuvre une meilleure représentation des moyennes et petites communes au sein des intercommunalités. Avec les critères qui s'appliquent aujourd'hui et à

La première a donné lieu à beaucoup de débats et n'a pas été retenue par le Sénat, qui a estimé qu'il existait un risque d'inconstitutionnalité- je le conteste, mais je comprends qu'on puisse le concevoir. En revanche, la seconde partie de cette proposition de loi a été logiquement reprise par nos rapporteurs et par la commission des lois- tout simplement parce qu'elle permet de favoriser l'accord local entre les maires, lorsque celui-ci est susceptible de permettre une meilleure représentation des petites et moyennes communes.

d'une disposition qui permet une véritable équité à l'égard des petites et moyennes communes, qui a été adoptée de manière très large par le Sénat

depuis fort longtemps, et plus précisément depuis la décision, qui a effectivement cassé un certain nombre d'accords locaux de représentation des communes au sein des conseils communautaires,

qu'il était loisible de déroger aux règles de répartition de droit commun pour cette métropole, définissant un régime dérogatoire qui aboutirait

provoquaient des écarts excessifs de représentation entre les communes membres, et que le régime dérogatoire- ce que nous appelons les accords locaux locaux -, dès lors que l'on prenait en compte cette représentation avec un écart de plus de 20 %, réduisait, au contraire, substantiellement et en moyenne, les écarts de représentation entre les communes. il nous semble que ce que la Constitution autorise, le législateur doit pouvoir le faire également, dans des conditions aussi rigoureuses. C'est pourquoi l'article que nous avons proposé, et que vous souhaitez supprimer, prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part des sièges s'écartant de ce fameux tunnel de plus ou moins 20 % à deux conditions cumulatives. Il faut tout d'abord que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation

qu'aucune commune ne doit se voir attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale. Voilà ce sur quoi s'appuie la proposition de la commission des lois.

absolument qu'un texte constitutionnel nous permette de donner cette profondeur. S'il n'y a pas de texte constitutionnel, ou si celui-ci était repoussé aux calendes grecques, je vous le dis, tout le travail que nous faisons aujourd'hui n'apporterait que des solutions s'apparentant

annoncée à plusieurs reprises et il a même adopté un texte en conseil des ministres, mais il ne saisit pas le Parlement, qui pourrait en délibérer et exprimer sa volonté. Les assemblées parlementaires ne peuvent exprimer d'autre volonté que celle qui résulte de leurs délibérations, à l'évidence. Si nous ne pouvons pas discuter d'une réforme constitutionnelle ayant de sérieuses chances d'aboutir dans un avenir immédiat, pourquoi ne saisirions-nous pas la chance de tenter d'aller explorer les marges de ce que le Conseil constitutionnel peut accepter pour favoriser une meilleure représentation des communes ? Au fond, la situation est simple, et ce n'est pas la peine de la décrire de manière complexe. Pour que chaque commune rurale, même faiblement peuplée, ait un représentant au conseil communautaire, il faut diminuer la représentation des communes intermédiaires de cette communauté de communes ; or celles-ci trouvent que c'est injuste, et elles ont raison. la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui limite la marge de manoeuvre des communes pour traiter cette question par des accords dérogatoires, est le reflet d'une vision trop étroite.

que les dispositions que nous avons adoptées pourraient être approuvées par le juge constitutionnel, à supposer qu'il en soit saisi. Je ne vois pas en quoi nous créerions une insécurité juridique en le faisant, puisque la loi, si elle passe après saisine devant le Conseil constitutionnel, ne comporterait pas de dispositions inconstitutionnelles, par hypothèse. Si le juge constitutionnel est saisi à l'occasion de l'application d'un accord il se prononcera sur la loi, mais tant qu'il n'y aura pas de raison de remettre en cause cet accord dérogatoire, il subsistera. il subsistera. Nous devons saisir la chance d'améliorer une situation avec bon sens et en respectant la liberté des élus et leur volonté commune, à laquelle le ministre nous a démontré qu'il était très attaché lui-même.

Sa jurisprudence n'est pas forcément figée. En outre, vous partez du principe que cette loi ne sera pas déférée au Conseil constitutionnel et que, par conséquent, avant sa promulgation, elle ne serait pas purgée

avoir l'audace de saisir le Parlement d'une réforme de la Constitution et, de l'autre, tenter raisonnablement, après un examen juridique approfondi, de faire évoluer les choses, je préfère de beaucoup la seconde solution, et c'est celle que je vous recommande. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

en amenant une plus juste représentation des communes et, soyons clairs, une plus juste représentation des petites communes, qui sont concernées au premier chef. Nous

transmis par le président de l'EPCI et à user plus régulièrement de la faculté d'audition de ce dernier devant le conseil municipal. La recommandation n° 10 consacrait, dans la charte de gouvernance de l'EPCI, un doit d'information et de participation de l'ensemble des conseillers municipaux sur les affaires intercommunales et prévoyait également les moyens nécessaires pour assurer sa pleine effectivité. Enfin, la recommandation n° 11 était de s'appuyer sur les réunions annuelles pour faire se rencontrer l'ensemble des acteurs de l'intercommunalité : conseillers communautaires, conseillers municipaux, directeurs de service, secrétaires de mairie et, parfois, partenaires sociaux. Nous avions même proposé, avec la recommandation n° 5, de conforter la capacité des conseillers municipaux membres des conseils communautaires à participer pleinement aux réunions, soit en recourant à la délocalisation des réunions, soit en s'appuyant plus systématiquement sur les technologies de type visioconférence, même si cela requiert un certain

les affaires intercommunales. C'est d'ailleurs un irritant, et même un urticant pour beaucoup d'élus. Cet article vise précisément à combler ce sentiment de déficit d'information des conseillers municipaux sur les affaires de leur EPCI. EPCI. Il consacre, d'une part, un droit à l'information sur les affaires faisant l'objet d'une délibération au sein de l'intercommunalité et prévoit, d'autre part, de les rendre destinataires de droit de la convocation et du compte rendu du conseil communautaire, ainsi que du rapport annuel sur les orientations budgétaires.

l'absence de réseau sur certains de nos territoires, et, d'autre part, au manque de maîtrise de l'outil informatique chez certains élus qui n'auraient pas encore reçu la formation nécessaire.

eu de formation spécifique. Enfin, il faudrait que chacune des communes réserve un espace pour l'affichage des informations concernant les délibérations des EPCI ou un registre dédié disponible pour l'information des citoyens en fonction des situations. L'article 4 vise à améliorer l'information des élus en leur adressant un certain nombre de documents relevant du fonctionnement des intercommunalités, que ce soit les convocations, les notes de synthèse, les comptes rendus. C'est une excellente disposition. En effet, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans les grandes intercommunalités, il existe un éloignement très préjudiciable entre les conseils municipaux et l'exécutif de l'intercommunalité.

Actuellement, cette note n'est envoyée qu'aux conseillers communautaires des EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus. Ce seuil ne nous paraît pas pertinent.

Conformément au code général des collectivités territoriales, le rapport annuel d'activité de l'EPCI fait l'objet d'une communication au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Avec la transmission des convocations, des comptes rendus et du rapport d'orientation budgétaire, les conseillers municipaux seront mieux informés sur les travaux de l'EPCI. Je propose d'élargir cette obligation de transmission au rapport annuel d'activité de l'EPCI, afin que les conseillers municipaux puissent préparer au mieux

d'avoir connaissance des décisions prises par le bureau communautaire. On le sait, la possibilité de délégation au bureau est assez large et n'exclut que les décisions ayant trait à l'ensemble des questions budgétaires. Autant dire que nombre de bureaux communautaires prennent la majeure partie des décisions importantes de leur intercommunalité. Ne pas transmettre l'information correspondant à ces décisions constituerait un manque de transparence.

communautaires ne peut matériellement pas être respectée immédiatement après l'installation des équipes issues du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.

Pour cette raison, le présent amendement vise à rendre facultatif cet envoi dans les trois premiers mois suivant l'élection du président de l'intercommunalité. Par ailleurs, le présent article prévoit que, si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. La mise en oeuvre de cette possibilité réduirait, dans la pratique, les délais d'envoi pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, elle impliquerait que ce dernier adresse plus en amont les documents à la commune, de façon que celle-ci puisse les envoyer à temps aux élus.

entre l'EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Quel

par l'EPCI ou par la commune membre si elle en fait la demande. Nous souhaitons rappeler que le Défenseur des droits a récemment fait savoir qu'il restait 541 communes classées en zone blanche, sans parler de celles où le haut débit n'est pas encore au rendez-vous. C'est pourquoi nous préconisons que ces documents soient consultables en mairie pour les conseillers municipaux qui en feraient la demande.

Cet amendement a pour objet de prévoir que le maire expose en séance du conseil, une fois par trimestre, les principaux sujets donnant lieu à délibération du conseil communautaire et la teneur des débats au sein de l'intercommunalité.

objet. En premier lieu, pour les communes de moins de 3 500 habitants, il tend à ajouter à l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal la transmission de l'ordre du jour et, plus important, d'une note de synthèse explicative sur les affaires soumises à délibération.

ceux d'opposition, l'ensemble des documents administratifs réglementaires préparatoires aux délibérations. Cette information préalable devrait permettre d'améliorer sensiblement la qualité des échanges et de la démocratie communale lors des conseils municipaux.

Par parallélisme des formes, nous proposons d'appliquer ce droit d'information à l'échelle du conseil municipal. Dans un souci de transparence et de bonne information de tous les membres du conseil municipal,

Je propose donc de préciser le contenu du rapport annuel d'activité de l'EPCI en y incluant le détail des actions par commune membre, pour chaque compétence, en matière de fonctionnement et d'investissement.

Avec cette proposition, j'ai bien conscience d'aller à rebours de l'esprit de ce texte de simplification. Cependant, je considère que ces EPCI disposent des moyens humains et financiers pour assumer cette tâche et que les rapports d'activité ne doivent pas

annuel d'activité, en y intégrant une présentation commune par commune de toutes les opérations réalisées, pour chaque compétence, en matière de fonctionnement et d'investissement, ainsi que de leur coût et des partenaires financiers concernés. Cette information est

Je propose de simplifier l'organisation des conseils municipaux en supprimant l'obligation, pour les représentants de la commune à l'EPCI, de rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI. En effet, les conseillers municipaux ont la possibilité d'interroger les représentants de la commune à l'EPCI lors de tout conseil municipal, sans qu'une disposition législative soit nécessaire

Ainsi, l'EPCI peut être amené à consulter les électeurs des communes membres sur les décisions que l'organe délibérant ou son président sont appelés à prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. À l'occasion de cette consultation, l'EPCI doit constituer un dossier d'information sur l'objet de la consultation, qui est mis à la disposition du public sur place au siège de l'EPCI et dans chaque mairie. Même si l'accès du public au dossier est assuré dans des conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, je propose de prévoir expressément la mise en ligne de ce rapport sur les sites internet de l'EPCI et des communes membres. Je propose également de préciser le contenu de ce dossier d'information, afin que les électeurs soient informés au mieux avant la consultation.

qui a été fragilisé, voire polytraumatisé, au fur et à mesure des différentes réformes territoriales. Nous avons tous été amenés à faire ce constat : chaque nouveau transfert forcé de compétences issu de la loi NOTRe a été un facteur de déstabilisation et, parfois, de démobilisation. L'article 5 A est important.

tout en visant la neutralité financière des restitutions de compétences aux communes. Cet article peut donc contribuer à débloquer des situations intercommunales tendues et à favoriser l'exercice d'une liberté locale au moyen d'un accord entre les parties.

définition limité par comparaison avec celui des compétences structurantes que sont les compétences obligatoires et les compétences optionnelles. Je pense que la suppression des compétences optionnelles est une hérésie

conséquence de la diminution de son coefficient d'intégration fiscale, sera compensée à due concurrence par une dotation de consolidation répartie entre ses communes membres au prorata de leur population dite « DGF ». Le droit actuel nous paraît pourtant clair en matière de transfert ou de restitution de compétences, puisqu'il dispose que les attributions de compensation doivent être modifiées après intervention de la commission locale d'évaluation des charges transférées lorsque l'EPCI à fiscalité propre à fiscalité propre est doté de la fiscalité professionnelle unique. Lorsqu'il est soumis au régime de la fiscalité additionnelle, les élus sont amenés à revoir les taux d'imposition communaux et intercommunaux en conséquence. Le financement des transferts ou restitutions de compétences est donc déjà assuré. Pour sa part, la dotation d'intercommunalité n'a jamais eu pour objet de financer l'exercice des compétences transférées à l'EPCI à fiscalité propre. Elle visait à encourager le développement de politiques publiques intercommunales supplémentaires,

Merci,

que l'EPCI continuera d'exercer les compétences optionnelles s'il les exerçait déjà, sauf si le conseil communautaire et les conseils municipaux décident la restitution aux communes des anciennes compétences optionnelles

réellement leur souhait de récupérer une compétence auparavant optionnelle, puisqu'une absence de délibération est considérée comme un avis favorable. Nous préférons que les communes puissent manifester leur volonté de récupérer une compétence devenue facultative

Cet article repose la question du transfert des compétences eau et assainissement, dont nous avons maintes fois débattu dans cet hémicycle et sur laquelle ma position est constante. Je plaide pour un retour au caractère optionnel de ces compétences,

conserver un caractère obligatoire. J'y vois une méconnaissance de ce que les élus locaux sont parvenus à mettre en oeuvre, souvent au prix de nombreuses heures de disponibilité et de travail bénévole, pour que les services de l'eau et de l'assainissement soient rendus de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible. Je rencontre les élus et les maires au quotidien dans la Drôme. Pouvoir conserver la maîtrise communale des compétences eau et assainissement eux une préoccupation constante et majeure. Contrairement à ce que j'ai souvent entendu dire, la grande majorité des investissements a été réalisée dans ces domaines par les communes, y compris les plus petites d'entre elles, avec le soutien des départements et des agences de l'eau. C'est le cas dans la Drôme, comme en témoignent les inaugurations fréquentes de stations d'épuration ou les opérations de rénovation des réseaux et des captages. Les élus locaux, je vous l'assure, ont un grand souci de la qualité du service rendu et de l'environnement. Le fait que ces compétences soient optionnelles n'empêche pas, et n'a d'ailleurs jamais empêché, les communes qui le souhaitent de les transférer, en tenant toujours compte de l'intérêt général et des besoins du service public. Je persiste donc à penser que la loi doit laisser les élus communaux décider eux-mêmes quelle est la meilleure solution. Laissons les territoires décider

relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Un pouvoir d'opposition au transfert est ouvert aux communes membres qui n'exercent pas ces compétences ou à l'une d'entre elles, à titre optionnel ou facultatif. Si 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale s'opposent, par délibération avant le 1 juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, la minorité de blocage est activée et le transfert reporté au 1 janvier 2026. Ce mécanisme de blocage vaut aussi pour les communes membres des communautés de communes qui exercent à titre facultatif un service public d'assainissement non collectif, ou Spanc. Conformément aux amendements déposés par le groupe socialiste lors de l'examen de la loi du 3 août 2018, repris par le présent projet de loi, cet amendement vise à élargir le pouvoir d'opposition des communes

mais il nous semble indispensable de permettre aux nouvelles municipalités qui seront élues en mars 2020 de s'exprimer sur ce sujet important.

de faire en sorte que la compétence eau redevienne facultative, c'est que, plus encore que la compétence assainissement, elle a un caractère tout à fait singulier. Nous sommes d'accord sur le constat, monsieur le ministre. Dès lors,

et propose désormais de supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Cette modification permettra ainsi aux communes n'ayant pas réalisé ce transfert de conserver ces compétences. Elles pourront toujours être transférées à l'avenir, sur la base d'une décision des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions de majorité habituelle. Néanmoins, il convient de préciser qu'une telle procédure peut s'accompagner, dans certains cas, de mauvaises surprises pour les EPCI. En effet, il arrive que des établissements publics soient amenés à prendre en charge un réseau communal dont ils ne connaissaient Cet amendement prévoit donc qu'un état des lieux, dont le contenu sera précisé par décret, soit fait par la commune en amont de la décision de transfert et transmis à la communauté de communes ou d'agglomération. Cette mesure de bon sens répond à un principe de transparence. Elle est demandée par de nombreux maires. L'amendement n° 680 rectifié

lors de réunions de présentation, des agences de l'eau ont fait savoir à des maires que les intercommunalités seraient désormais prioritaires pour l'attribution des subventions, ce qui ne laisserait qu'un hypothétique reliquat pour les communes ayant conservé les compétences. Il s'agit là d'une pression supplémentaire exercée sur les maires,

aux communautés de communes et d'agglomération, ainsi que de la catégorie des compétences optionnelles. Nous proposons de le compléter en supprimant les compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles

obligatoire- aux intercommunalités à 2026 si « au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population » le souhaitent. Cela n'a rien changé aux problèmes de fond soulevés par les élus. Ce transfert retire une nouvelle compétence aux maires, et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles aux communes. Il contraint à des regroupements de services qui n'avaient pas, jusqu'à présent, le même mode de gestion.

le précédent. La coopération en matière d'eau et d'assainissement est bien antérieure à la coopération intercommunale, puisque les syndicats d'alimentation en eau potable existent depuis longtemps. Leur périmètre dépasse les limites des territoires, des agglomérations, des EPCI, des départements, voire des régions. Il est donc davantage lié à la géographie naturelle qu'à la géographie administrative. La nature du territoire ne dépendant pas du statut de l'EPCI, dans certaines communautés urbaines, voire certaines métropoles, les surfaces agricoles ou rurales sont plus importantes que les superficies réellement urbanisées, notamment du fait de la constitution d'EPCI « XXL

qui, contrairement à ce qui est parfois interprété, traduit une situation de dépendance en termes de flux de déplacements commerciaux, mais ne caractérise pas la nature physique du territoire, et donc n'intègre pas les contraintes et les facteurs de pertinence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement.

D'un côté, le Gouvernement nous propose de revoir une nouvelle fois les possibilités de blocage de ce transfert, en se contentant de les reporter et de créer un dispositif complexe de délégation qui ajoute peu aux possibilités actuelles, voire les restreint. D'un autre côté, la commission des lois va plus loin et propose de supprimer le transfert obligatoire aux communautés de communes et d'agglomération. Cette mesure a le mérite d'être limpide, mais elle ne suffit pas.

Lutter contre la différenciation territoriale des EPCI pour la répartition des compétences permet aussi de lutter contre certains effets pervers de la gestion de l'eau et de l'assainissement.

Pour offrir une solution à toutes les communes, il faut rendre les compétences eau et assainissement facultatives pour tous les types d'EPCI.

14,6 premiers mètres cubes par année et par personne, soit 40 litres par jour. Le droit à l'eau est clairement défini en droit positif, notamment depuis l'adoption sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Le droit humain d'accès à l'eau potable, l'assainissement et à l'hygiène fait également partie des dix-sept objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies en août 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d'eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d'hygiène de base. Afin de rendre effectif ce droit, qui demeure aujourd'hui largement fictif, nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d'eau par jour,

la gratuité n'est pas le produit débarrassé du coût, mais bien du prix ! Ce dernier n'est donc pas le problème de l'usager, il redevient un élément dans le cadre de la gestion d'un service public industriel et commercial, soit un coût pour le gestionnaire.

Ce droit, inscrit dans le code de l'environnement, concerne potentiellement 2 millions d'habitants pour lesquels la facture d'eau et d'assainissement dépasse le seuil d'acceptabilité, soit 3 % du revenu.

je citerai Henri Emmanuelli, qui disait : « Notre société doit garantir à tous un accès à l'eau potable et à l'assainissement- cela fait écho, madame Assassi, à vos propos. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun qu'il convient de préserver. de préserver. Sa gestion dans le cadre du service public demeure fondamentale. » Elle est fondamentale, parce que l'impact sur le prix n'est bien entendu pas le même, ce qui explique une partie de nos préventions à l'égard de telle ou telle privatisation, suivez mon regard Dans son discours d'août 2018, aux Assises de l'eau, le Premier ministre a rappelé la volonté du Gouvernement d'accélérer le déploiement de la tarification sociale de l'eau. Il s'agit, monsieur le ministre, de la mesure 17 de ces assises Le Gouvernement souhaite voir se généraliser la tarification sociale à destination des populations les plus fragiles. » Il faut donc une offre nouvelle aux collectivités volontaires, et on leur propose de mettre en place le chèque eau, sur le même modèle que le chèque énergie. Le Gouvernement entend donc bien faire de la tarification sociale de l'eau une politique publique Si l'amendement présenté par le Gouvernement vise à généraliser le dispositif de la tarification sociale de l'eau- nous nous sommes ralliés à sa rédaction -, il tend pourtant à faire porter l'intégralité du dispositif

Par-delà, il s'agit de véritables enjeux sociaux et écologiques. L'eau constitue un véritable poste de dépense pour le budget des ménages. Il est donc intéressant de permettre la mise en oeuvre de ce droit inaliénable et universel d'accès à l'eau. L'adoption de cet

Cette tarification sociale s'inscrit dans les objectifs de développement durable, les fameux ODD, qui sont au nombre de 17. Elle correspond plus exactement à l'objectif n° 6. Ces ODD forment l'essentiel de l'agenda 2030 et sont complémentaires de l'accord de Paris sur le climat, qui nous engage collectivement.

Aujourd'hui, en France, la moitié des eaux de surface ne sont plus potables. Cette dégradation s'explique par la présence de pesticides, de métaux, de mercure, de déchets médicamenteux et autres molécules artificielles non dégradables naturellement, sans oublier les micro-plastiques et les nano-plastiques, que nous commençons à découvrir.

politique de sensibilisation et d'incitation, afin de réduire les prélèvements sur la ressource en eau. Des expériences le prouvent de manière non négligeable moins on consomme d'eau, moins l'eau est chère. Cela a permis une baisse générale de la consommation, notamment à Dunkerque. La prise de conscience par chacun de son empreinte eau et l'adoption d'un comportement responsable sont au coeur de cet amendement. Ce dernier, par ses fins écologiques, est absolument nécessaire dans le contexte actuel. Ce n'est plus à démontrer : il est grand temps de permettre ces dispositifs, qui sont propres à créer du progrès, de la solidarité et de l'écologie. La parole

insistait sur la volonté du Gouvernement d'accélérer le déploiement de la tarification sociale de l'eau. J'ai donc regretté qu'elle n'apparaisse plus dans la version présentée en conseil des ministres, alors qu'elle figurait dans l'avant-projet. J'ai souhaité que ce débat fasse partie des travaux de la commission, mais malheureusement l'amendement du RDSE a été frappé d'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. Je salue donc votre démarche, monsieur le ministre, de généraliser une expérimentation permise dans la loi Brottes. Elle prévoit que les services publics de l'eau et de l'assainissement soient autorisés à mettre en oeuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous, ainsi que cela est prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Conformément à ce que nous avions proposé, cette aide pourra prendre la forme de versements d'aides ou de tarifs progressifs dans la tarification de l'eau,

d'un amendement d'appel. Les communes et les maires souhaitent que l'on cesse de transférer des compétences qui les dépouillent de leur pouvoir dans différents domaines, notamment en matière d'urbanisme. Même si l'on peut avoir une conception intercommunale de l'urbanisme, il importe de

Or c'est encore la commune qui supporte la retenue financière pour manque de logements sociaux, et c'est le maire qui a la responsabilité d'assurer la tranquillité publique de ses concitoyens au titre du pouvoir de police. Le maire est en

Gouvernement ? La mort est une chose suffisamment sérieuse pour que le Gouvernement y prête une attention toute particulière. Dans la relation que nos concitoyens peuvent avoir avec les autorités locales,